demande de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et du groupe Les Républicains, sur l'avenir de l'audiovisuel public. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. que les orateurs de la commission et du groupe qui ont demandé ce débat disposeront d'un temps de parole de dix minutes, y compris la réplique, puis le Gouvernement répondra pour une durée équivalente.

Monsieur le président, madame la ministre, mes très chers collègues, face à la mutation numérique, je me suis attachée de longue date à ce que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication réfléchisse et travaille, en lien avec la commission des finances, à l'avenir de l'audiovisuel. Ainsi, il y a bientôt trois ans, était engagé au Sénat le débat sur une profonde réforme de l'audiovisuel public à l'occasion de la publication du rapport de nos collègues, que je salue, Jean-Pierre Leleux et André Gattolin. Les recommandations de ce rapport demeurent très largement d'actualité. nous avions sans doute encore sous-estimé l'ampleur de la révolution technologique en cours qui menace jusqu'à la pérennité d'un secteur audiovisuel, privé comme public d'ailleurs, exposé aux coups de boutoir de la concurrence des grandes plateformes américaines, bouleversant totalement nos usages et nos modèles économiques. Nous sommes, en fait, face à une situation que l'on pourrait résumer ainsi : l'audiovisuel public est-il encore capable de répondre aux attentes de tous ses publics, notamment des plus jeunes, qui ont accès à des milliers de programmes sur des plateformes numériques ? Les programmes publics se distinguent-ils suffisamment des programmes privés- par leur audace, leur spécificité, leur qualité -pour justifier un financement public à hauteur de 3,7 milliards d'euros ? Ces entreprises publiques ont-elles bien pris la mesure des évolutions en cours et sont-elles prêtes à changer de logiciel pour relever le défi, ce qui implique nécessairement de modifier certaines habitudes ? Autant le dire tout de suite, la réponse à ces trois questions est loin d'être évidente ! Les plus jeunes de nos concitoyens ne regardent plus la télévision publique, dont les téléspectateurs ont largement dépassé la moyenne d'âge de soixante Ses programmes sont considérés comme peu innovants et peu exportables. Quant à la situation financière de ces entreprises, il faut distinguer Arte, France Médias Monde et l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, qui font des efforts pour contrôler leurs dépenses, de France Télévisions et Radio France, dont les coûts de structure poursuivent, malgré les efforts, leur progression, notamment quant à la masse salariale. Au-delà des missions à redéfinir, c'est aussi le financement de ces entreprises qui pose question.

par les plateformes numériques et ne peut donc constituer une ressource d'avenir. Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public, la CAP, reste fondé sur la possession d'un téléviseur. Or le taux d'équipement baisse à mesure que progressent les nouveaux usages sur les supports numériques. Une réforme de la CAP est donc devenue indispensable. nous devons faire un choix. Soit l'audiovisuel public- notamment France Télévisions -poursuit sur la pente de la banalisation de son offre, et c'est la légitimité même d'un financement public qui pourrait être- tôt ou tard -posée. Soit on estime que cet audiovisuel public a un rôle à jouer en termes de culture, d'éducation et de démocratie- ce que je crois profondément -, et alors il faut mettre en oeuvre une réforme systémique. Ce choix de société doit concerner tous les Français. C'est pourquoi nous sommes heureux d'ouvrir aujourd'hui, en votre présence, madame la ministre, ce grand débat d'intérêt national. Autant le reconnaître, il n'y a pas d'unanimité pour défendre le service public Il y a ceux qui ne jurent que par la course à l'audience et à la publicité, pour le privé comme pour le public. Il y a ceux qui estiment que l'audiovisuel public coûtera toujours trop cher et qu'il faut réduire ses moyens. Il y a ceux, de moins en moins nombreux, qui jugent qu'il ne faut rien changer et qu'il faut continuer à augmenter les dépenses de l'audiovisuel public. Il y a enfin, et c'est nouveau, toute une partie de la population qui considère qu'elle ne doit payer que ce qu'elle consomme et refuse donc- par principe -d'acquitter une redevance. Ce débat, nos voisins suisses sont en train de le conduire,

Face à cette menace, la SSR a pris acte de la nécessité de se transformer avec un maître mot : rendre accessible l'ensemble des contenus télévisés et radiophoniques sur une plateforme globale multisupport et renforcer l'attractivité de ses programmes.

Renforcer la spécificité de l'audiovisuel public ; donner la priorité à l'audace, à l'innovation, à la rigueur ; regrouper l'ensemble des programmes sur une même plateforme numérique ; opérer des mutualisations de services par thématique- information, culture, sport, territoires : telle doit être notre ambition. Nous devons aller jusqu'au bout de la révolution des usages et ne pas nous apitoyer sur des structures qui nous sont, certes, familières, mais qui sont vouées à se transformer radicalement si elles veulent perdurer. D'ici peu, les téléspectateurs regarderont d'abord leurs programmes de manière complètement délinéarisée et sur internet à travers les télévisions connectées. Pour la radio, on peut penser que la 5G attendue pour 2020 constituera également une nouvelle frontière permettant de dépasser l'antique FM et ses problèmes de pénurie de fréquences. Le changement de paradigme technologique emporte la nécessité de repenser l'organisation des sociétés de l'audiovisuel public et, donc, de leur gouvernance. La commission continue de penser que la création d'une permettrait d'assurer la coordination des moyens et le développement d'une offre nouvelle dans le respect des identités des entreprises et des personnels. Nous n'avons jamais proposé de fusion, car cette forme de rapprochement aurait aussi un coût social important, dont il appartient au Gouvernement de mesurer l'ampleur. C'est l'option qui a été privilégiée par nos voisins suisses, belges et britanniques, mais elle comporte le risque d'y laisser beaucoup de temps et d'énergie, au détriment d'une mise en oeuvre rapide des adaptations nécessaires. Ce qui importe- au-delà des systèmes et des schémas de rapprochement -, c'est de permettre aux salariés de ces sociétés de retrouver confiance dans l'avenir de l'audiovisuel public. Pour cela, soyons pragmatiques L'audiovisuel public a besoin d'être incarné par une personnalité dont la mission consistera à garantir, devant la Nation, l'indépendance de l'institution, la déontologie de l'information, le respect du pluralisme et l'équité de la répartition des crédits issus de la CAP entre les différentes entreprises, sans préjudice notamment pour la chaîne franco-allemande Arte et l'audiovisuel extérieur, qui font un travail remarquable. À cet égard, je déplore, au regard des responsabilités de la présidente de France Médias Monde, l'absence de discernement qui a mis un terme de manière mécanique à son mandat. Compte tenu de cette ambition, nous devons trouver un mode de nomination indiscutable, sachant que tout ou presque a été essayé dans ce domaine, sans donner satisfaction. Un consensus semble se dessiner pour prévoir une nomination par le conseil d'administration. Il va de soi que cette modalité de nomination n'aura de sens que si l'indépendance des membres du conseil d'administration est garantie, ce qui signifie que la représentation des tutelles soit simplifiée. Des missions réaffirmées, une ambition culturelle et éducative renforcée, des personnels remobilisés, une gouvernance commune et indépendante instaurée, ces piliers de la réforme doivent être consolidés par une profonde modernisation de la contribution à l'audiovisuel public pour garantir, dans la durée, les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions. Là encore, la proposition formulée par nos collègues Jean-Pierre Leleux et André Gattolin, en 2015, d'une contribution forfaitaire universelle sur le modèle allemand apparaît comme le chemin le plus solide pour boucler cette réforme systémique. Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons penser cette réforme pour les quinze ou vingt années à venir. En toute logique, nous devons également nous interroger sur l'adaptation de la régulation au nouveau contexte marqué par le numérique.

il nous faut conduire ce travail. Avec le développement de la réception par la fibre, l'avenir de la télévision numérique terrestre, la TNT, est également en jeu, et donc la réglementation imposée aux grandes chaînes qui repose sur l'attribution d'une licence de diffusion hertzienne. Une simplification de cette réglementation constitue un horizon sans doute incontournable pour permettre un développement de la production française, notamment à l'export. Il en est de même, madame la ministre, de la chronologie des médias, qui a besoin d'être modernisée. Nous avons fait des propositions en juillet dernier pour favoriser les comportements vertueux de ceux qui investissent dans le cinéma. Nous souhaitons qu'un accord soit trouvé, faute de quoi le législateur devra tirer les conséquences de cette situation. On le voit, tous ces changements sont liés. C'est donc à une réforme globale qu'il faut penser. Comme je vous l'ai écrit, madame la ministre, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication est prête et compte jouer tout son rôle dans le débat qui va s'engager à partir de maintenant. Nous poursuivons d'ailleurs nos travaux et nous engagerons très prochainement un travail de fond sur France 3 et France Bleu, les chaînes des territoires, et sur bien d'autres sujets encore.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, jamais le choix du téléspectateur-auditeur-citoyen n'a été aussi varié et aussi large qu'aujourd'hui, et cette diversité de choix devrait se renforcer encore sous l'effet de la concurrence et de l'arrivée de nouveaux acteurs issus du numérique. En France même, il y a cinq chaînes d'information continue, plusieurs chaînes consacrées au sport- gratuites et payantes -, une multitude de chaînes dédiées au cinéma et à la production audiovisuelle, aux séries, des chaînes de musique, et la même diversité s'observe sur les ondes radiophoniques. ces conditions, quelles sont les justifications de l'existence d'un audiovisuel public qui bénéficie chaque année de plus de 3,7 milliards d'euros de fonds publics et de 400 millions d'euros de recettes publicitaires ? La question se pose, en effet, et nous l'entendons de-ci, de-là. Pour ma part, et je partage avec la commission de la culture cette idée forte, j'ai la conviction qu'un audiovisuel public puissant est nécessaire, pour autant que son offre soit différenciée et qu'il joue un rôle de référence, en particulier dans l'information et l'accès à la culture. L'explosion des offres audiovisuelles, le développement des réseaux sociaux exigent, de mon point de vue, la présence d'un axe public fort qui se distingue dans le paysage global de l'audiovisuel ; nous y reviendrons. L'existence d'un pôle audiovisuel extérieur puissant est une nécessité. C'est la vision de la France dans le monde, même si on peut parfois s'interroger sur l'intérêt que des fonds publics financent des programmes en langue anglaise. Voilà sans doute une piste de réflexion sur des économies ou des redéploiements possibles. Mais France Médias Monde, qui, dans ce système-là, n'a que peu de valeur ajoutée par rapport à la BBC et à CNN, fait un travail remarquable pour l'image de la France à l'extérieur. Les programmes de Radio France sont, pour l'essentiel, conformes aux attentes, même si des doublons peuvent exister avec certaines offres privées, ainsi entre France Musique et Radio Classique. Le bilan de la chaîne franco-allemande Arte est, pour sa part, conforme au projet de ses concepteurs : ouverture culturelle et internationale, exigence et accessibilité des programmes, invitation à la curiosité et à la découverte, ambition européenne. L'enjeu principal est donc double. Il est temps, tout d'abord, de redéfinir les missions de France Télévisions, qui a aujourd'hui une double identité, à la fois publique et commerciale. Il faudra lever cette ambiguïté ; c'est le rôle du législateur. Depuis des années, l'absence de décision sur ce sujet a compliqué la gouvernance et la gestion du groupe. sommes convaincus que rien ne justifie de payer une redevance annuelle de 139 euros pour des programmes souvent disponibles gratuitement sur les chaînes privées. Rien ne justifie, non plus, de conserver des programmes aussi coûteux

Il nous revient, enfin, de nous interroger sur l'usage qui est fait des 400 millions d'euros consacrés chaque année à la production audiovisuelle, compte tenu du caractère peu innovant et insuffisamment marquant des programmes ainsi financés. Le second enjeu concerne la transition numérique, qui doit nous conduire à nous interroger. Le contribuable est en droit d'accéder à tous les programmes du service public sur une même plateforme accessible sur tous les supports, ce qui nécessiterait un regroupement des contenus produits par les différentes sociétés de l'audiovisuel public.

coûteuse à développer, sans proposer une offre vraiment distincte. Que faut-il penser de ce projet, qui a d'ailleurs pris beaucoup de retard ? Madame la ministre, nous souhaitons que l'avenir de l'audiovisuel public passe par une clarification de ses missions, de son périmètre et de ses projets. public n'a ni les moyens financiers ni les compétences technologiques pour concurrencer une grande part du privé dans le paysage médiatique qui s'annonce. Il doit tracer une voie complémentaire, avec des exigences et des moyens spécifiques, comme mon collègue André Gattolin Comment donner la priorité à la culture, à l'éducation, au débat démocratique, à la curiosité et à l'ouverture, tout en continuant de subir la pression de l'audimat et des recettes publicitaires ?

Les regroupements et la clarification des missions du service public de l'audiovisuel doivent permettre d'engager une nouvelle étape fondée sur la différenciation de son offre, un financement spécifique, à travers la réforme de la CAP et la recherche d'une qualité accessible à tous. La parole

Peut-être, madame la ministre, avant d'envisager une extension de cette redevance, devrait-on demander à l'audiovisuel public, au-delà des questions de gouvernance, de faire des économies de gestion. aux particuliers, aux collectivités, aux entreprises. Peut-être l'audiovisuel public, en se réorganisant, en veillant à ne pas encourir de dépenses excessives sur certains domaines, pourrait-il de même s'efforcer de rationaliser sa dépense.

on ne peut pas dire que, si l'on compare les coûts de production de l'ensemble des chaînes de télévision, il y ait toujours, du côté du service public, un plus par rapport aux chaînes privées.

Il fut un temps où il y en avait moins, et où l'on n'avait pas pour autant le sentiment que le service public était nul ou insuffisant. Fallait-il absolument créer, récemment,

l'extension de la redevance, avant de demander aux Français un effort supplémentaire pour l'audiovisuel public, peut-être peut-on demander à celui-ci de réformer ses méthodes de gestion,

trouver, peut-être, plus de rationalité. En attendant, madame la ministre, nous participerons volontiers à votre réflexion sur la réforme. Nous vous demanderons seulement de réfléchir avec l'ensemble des responsables aux moyens de réguler la dépense avant de déterminer s'il faut augmenter la recette.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie la commission de la culture et le groupe Les Républicains d'avoir sollicité ce débat de contrôle, qui me permet de rappeler le sens de la transformation que nous engageons dans l'audiovisuel public, de présenter la méthode que nous avons choisie pour avancer, et de vous faire un point d'étape sur nos réflexions.

La transformation de l'audiovisuel public est aujourd'hui incontournable. Plusieurs de nos voisins européens l'ont engagée, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention, madame la présidente de la commission. C'est pourquoi je me suis rendue à Londres afin de rencontrer les dirigeants de la BBC

Cinq chantiers ont d'ores et déjà été identifiés : la reconquête des jeunes publics, l'international, l'offre de proximité, l'offre en ligne et les synergies sur les ressources transverses.

Elle doit aussi pouvoir se nourrir des travaux parlementaires, qui sont particulièrement riches sur ce sujet. Je pense singulièrement aux travaux de votre commission, madame la présidente, travaux dont je salue la qualité. Je connais par ailleurs votre investissement personnel sur ces questions.

ce qui est du calendrier, comme nous l'avons déjà indiqué, nous ferons nos annonces d'ici à la fin du mois de mars.

eux, ce sont les contenus et les programmes. Nous touchons ici à la raison d'être de l'audiovisuel public : sa singularité et ses missions. Vous l'avez bien souligné

La question centrale est la suivante : comment continuer à faire la différence ? C'est véritablement la boussole de la transformation. Nous avons identifié plusieurs missions prioritaires : j'en évoquerai trois.

Il faut maintenant reconquérir les adolescents et les jeunes adultes, qui délaissent la télévision linéaire, mais consomment beaucoup de contenus en ligne et, notamment, de vidéo à la demande. Les deux tiers des 15-24 ans regardent des vidéos en ligne quotidiennement sur cinq est abonné à une offre de vidéo à la demande, contre une personne sur douze pour la moyenne de la population. L'audiovisuel public doit leur proposer, sur le canal numérique, une offre de contenus culturels, éducatifs et informatifs de référence que les jeunes ne trouveraient pas ailleurs. Une autre mission prioritaire de l'audiovisuel public la proximité. L'offre d'informations et de programmes locaux est une spécificité de l'audiovisuel public. Elle est fondamentale pour la vie de nos territoires ; ce n'est pas à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, que je l'apprendrai. Pour renforcer cette mission, je crois à une coopération accrue entre les antennes de France Bleu et France 3, afin de produire davantage d'émissions et de programmes locaux. Les équipes travaillent à des expérimentations, notamment autour d'une matinale.

Les efforts des sociétés sont aujourd'hui éparpillés ; il faut plus d'investissements et d'offres numériques communes. Les sociétés font à l'heure actuelle des propositions en ce sens. Il faudra aussi répondre, à terme, à l'enjeu du média global, qui mêle image, son et voix, et qui est présent en linéaire comme en non-linéaire. troisième enjeu de la transformation est la gouvernance de l'audiovisuel public. Nous avons une volonté claire : renforcer la coordination entre les différentes sociétés. Nous avons ouvert pour cela plusieurs pistes de réflexion.

simplement issue du parangonnage- pour ne pas dire du -que nous avons effectué auprès des modèles européens, notamment de la BBC. À ce stade, nous ne privilégions pas le meccano institutionnel consistant à créer une nouvelle entreprise unique. Nous préférons des méthodes souples d'organisation, qui favoriseraient la mise en oeuvre rapide des réformes. rapide des réformes. La question d'une nomination des dirigeants par les conseils d'administration se pose. Cette piste a été évoquée par le Président de la République pendant la campagne présidentielle. Elle donnerait aux dirigeants une plus grande assise managériale et impliquerait de revoir la composition des conseils d'administration. Les suggestions émises par le sénateur André Gattolin dans sa proposition de loi nous offrent une base de travail, qui sera complétée par d'autres propositions.

je l'ai réaffirmé lors de l'examen du budget pour 2018, il n'y aura pas de retour de la publicité après 20 heures sur France Télévisions. C'est un élément fort de distinction du service public. S'agissant de la redevance, comme je l'ai déjà dit, je souhaite qu'un débat soit ouvert. À moyen terme, l'évolution des usages pose la question du rendement de cette contribution et de l'équité entre contribuables. Nous aborderons la question sans tabou.

réflexion. Pour ma part, le rôle de régulateur du CSA ne me dérange pas : il faut bien qu'il y ait un organe régulateur. Ce qui pose problème, à mon sens, c'est que l'on donne à la même institution le pouvoir de nomination et le pouvoir de régulation.

enrichir culturellement le plus grand nombre par des programmes ambitieux en matière de création artistique et une démocratisation de l'accès à la culture. Cette volonté d'accès élargi de nos concitoyens à la culture

davantage de programmes culturels sur nos médias, notamment sur la télévision et la radio publiques. D'ailleurs, l'augmentation d'audience de certaines chaînes culturelles spécifiques constitue d'une certaine façon un indicateur de cette demande. Dans un récent sondage, les Français indiquaient qu'ils voudraient plus de films- presque à 70 % -, plus de culture- presque à 50 % -et plus de documentaires- à 48 % -sur France Télévisions. Il suffit de voir le tollé qu'a suscité l'idée de supprimer certains documentaires sur France Télévisions pour se rendre compte de l'attachement des Français à ces émissions. La culture est clairement identifiée

au secteur de la création. En effet, n'oublions pas que France Télévisions représente la moitié des investissements dans la création audiovisuelle française. L'offre culturelle est aussi identifiée comme un chantier où les coopérations

le débat s'organiserait déjà autour de vos conclusions, avant même qu'il se soit engagé dans le pays. En somme, nous proposons une méthode pluraliste et démocratique, qui fait appel à l'intelligence citoyenne. Je crois que le pays a beaucoup

je consulte beaucoup -, avec les gens sur le terrain- je me déplace : je me suis rendue à France 2 ou France 3 pour rencontrer les équipes -et avec le Parlement.

ce qui est de l'ordre de la responsabilité des pouvoirs publics dans un environnement concurrentiel, c'est plutôt de faire la promotion du service public, parce qu'il y a des concurrents, et non de faire preuve de dénigrement- tel n'a

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission de la culture, mes chers collègues, face à l'évolution des usages et des technologies, face à la concurrence des chaînes privées et aux nombreuses contraintes budgétaires, l'audiovisuel public, machine forte de 18 000 salariés et de 3,8 milliards d'euros de budget, s'essouffle, en termes tant de modèle que de contenus. Il nous faut le réinventer : il s'agit là d'un chantier d'ampleur, nous en convenons tous. Cependant, en élevant l'audiovisuel public français à la hauteur d'un service d'excellence, c'est l'image de la France qui se relèvera la France des territoires, la France nationale, la France à l'étranger. Pour cela, nous sommes d'accord, une réforme en profondeur est nécessaire. Sur la forme, il nous faut sans doute harmoniser la gouvernance, revoir le financement, mutualiser les moyens. Toutes ces questions sont essentielles. Avant tout, il est nécessaire d'adopter une vision claire des missions que le Gouvernement souhaite confier aux médias publics. Il nous faut redéfinir leur périmètre et définir leur raison d'être. On demande à l'audiovisuel public de remplir trois missions : éduquer, informer et distraire. Actuellement, ces missions se confondent en partie avec l'offre privée ; en partie seulement, car l'éducation citoyenne reste l'apanage du service public. À l'heure de la désinformation, redonnons une pleine dimension à cette mission d'éducation à la fois citoyenne et populaire. À cette mission originelle, ajoutons celle du rayonnement de la France dans le monde francophone. Faisons de l'audiovisuel public le premier vecteur d'identité et de cohésion nationale sur nos territoires et à l'étranger.

L'audiovisuel public a un rôle décisif à jouer dans ce domaine, j'en suis convaincue. D'ores et déjà, des initiatives sont menées sur les antennes avec des programmes de décryptage et de vérification, par exemple sur

en Grande-Bretagne, 85 % des jeunes révisent en utilisant la BBC comme support d'information

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie ou encore le Qatar s'étaient auparavant dotés de canaux semblables. Même si les programmes de France 24 n'ont pas prioritairement vocation à être diffusés dans notre pays, il me semble opportun de leur offrir une véritable visibilité nationale,

ensuite de rendre plus acceptable la contribution, par l'impôt, des citoyens au service public audiovisuel. Il nous paraît souhaitable, voire logique, que celles et ceux qui financent la chaîne de la France à vocation internationale puissent y accéder plus largement. faire pour la qualité des programmes diffusés par France 24. Alors que les sujets internationaux sont, à mon sens, « sous-traités » dans la plupart des médias d'information télévisuels, cette chaîne représente une source d'information précieuse pour nos concitoyens. À l'heure de la mondialisation, porter un regard éclairé au-delà de nos frontières ne semble pas superflu. En outre, l'actualité ne se résume pas à une succession de faits divers ou à la phrase politique assassine du jour. France 24 est désormais accessible depuis la TNT, soit aux seuls Franciliens, soit entre minuit et six heures du matin lorsque France Info TV interrompt ses programmes. Madame la ministre, nous sommes nombreux à regretter que cette visibilité ne soit pas encore plus grande. Pouvez-vous nous dire si l'offre de France 24, assez complémentaire de l'offre d'informations télévisuelles aujourd'hui proposée, a selon vous vocation à être plus aisément accessible sur le territoire national ? La parole

l'audiovisuel public est avant tout un service public. C'est pourquoi le futur projet de loi doit d'abord être projet de loi d'orientation, permettant de clarifier les missions qui lui sont dévolues. Une fois ces missions précisées, il sera temps de réfléchir aux moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qui auront été fixés. Pour parvenir à ce résultat, une réflexion et un débat ouvert sont nécessaires. Un projet partagé est en effet un projet accepté et, souvent, plus facile à financer.

j'aimerais insister sur le défi majeur que représente l'éducation des jeunes à l'audiovisuel public. À l'heure où les plus jeunes se désintéressent de nos médias nationaux et sont exposés quotidiennement à des, il faut parvenir à cultiver, divertir et informer notre jeunesse avec des programmes de qualité conçus pour elle, afin que nos enfants se réconcilient avec l'audiovisuel public et prennent l'habitude de l'utiliser. Pour y arriver, il faudra aussi se poser la question de la forme des programmes, avec le développement des formats digitaux, de la présence sur les réseaux sociaux, ou encore de l'opportunité de fusionner l'ensemble de ces programmes sur une seule chaîne consacrée à la jeunesse. La parole

durablement s'éloigner du public jeune. L'un de nos paris est d'accompagner cette transformation pour qu'il soit à nouveau en mesure de proposer des programmes attractifs de façon linéaire ou délinéarisée, correspondant aux usages des jeunes et prenant véritablement en compte la problématique de ces Des pistes sont déjà en cours. Je pense, notamment en matière d'offre, au Mouv'ou à cette toute nouvelle plateforme que France Télévisions vient de lancer, Slash,

Nous sommes nombreux à penser que, depuis trop longtemps, l'audiovisuel public français se situe bien trop loin des aspirations du public et qu'une restructuration en profondeur est absolument nécessaire. Face à ce qu'il convient d'appeler « une crise du financement », il est devenu indispensable de refonder un nouveau modèle qui permettra de garantir des ressources dans la durée, de clarifier le rôle de l'État et de renforcer la cohérence de l'audiovisuel public. Ce nouveau modèle doit permettre de concilier une meilleure maîtrise des ressources de l'audiovisuel public et de ses dépenses, avec la nécessité de dégager des marges de manoeuvre, notamment afin d'améliorer son offre numérique. avant de parler des moyens, il semble indispensable de réaliser un véritable audit de l'ensemble, un audit sérieux, financièrement analytique, afin de pouvoir identifier de façon certaine et transparente les coûts réels, aujourd'hui noyés dans un ensemble opaque. un ensemble opaque. Périmètre d'intervention incertain, gestion pléthorique des ressources humaines, retard pris dans le développement du numérique et sa marginalisation dans la maison, filière dispendieuse du service de production interne : c'est un euphémisme de dire qu'une rationalisation est souhaitable. Que dire des personnels, indiscutablement de bonne volonté dans leur grande majorité, mais qui, par manque de considération, ont peur du changement ? Où en est, par exemple, l'accès à la formation ? Où en est la fameuse GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ? Où en est l'audit social, technologique et financier nécessaire à la compréhension de l'ensemble de l'audiovisuel public français et sur lequel s'était engagée Mme Ernotte, présidente de France Télévisions ? Alors, madame la ministre, mes chers collègues, si une restructuration en profondeur est aujourd'hui absolument nécessaire, elle n'est possible que si des objectifs clairs sont fixés.

parlez de gestion des personnes, de transformation, etc. Or un des points importants sur lesquels nous avons insisté dans ces comités stratégiques, et qui correspond d'ailleurs au travail sur les synergies possibles de coopération, c'est la formation c'est la formation des personnes. L'audiovisuel public se transforme. Si l'on se contente de le regarder se transformer, la catastrophe est certaine. Si l'on essaye d'accompagner cette transformation,

pour le journal de France 3. Au passage, ce changement d'habillage était programmé dès 2017, mais, à l'heure des négociations budgétaires, on avait un peu de mal à justifier un tel changement : changer l'habillage et l'identité suppose de profonds changements à l'antenne, ce qui n'était pas le cas. Ces choix cosmétiques, qui ont des incidences budgétaires dont on ne connaît d'ailleurs

à la veille de la préparation d'une nouvelle grande réforme. Il a été décidé de changer de stratégie : après un retour à la verticalisation et à l'organisation par chaînes séparées- France 2, France 3 et les autres chaînes -, on en revient à l'idée de la création soudaine d'une organisation organisation transverse, telle qu'elle avait d'ailleurs été envisagée au moment de l'entreprise unique sous la présidence de Carolis. On se retrouve là face à un projet qui est exactement le contraire

Monsieur le sénateur, vous êtes au courant de l'indépendance totale des médias et de l'audiovisuel public !

amener de la culture -, il faut repenser l'audiovisuel public au regard de tous les chiffres que nous avons partagés, en tenant compte de la nécessité de rendre les choses beaucoup plus lisibles et d'être attentifs

toucher les jeunes, tout en se préoccupant aussi des Français éloignés- on parle beaucoup du numérique, mais il ne faut pas oublier que 30

Les citoyennes et les citoyens de ce pays ont besoin d'informations de qualité, de débats contradictoires, de mises en perspective historiques et philosophiques. Le meilleur antidote contre les « fausses nouvelles »- je le dis en français c'est la connaissance, dans la mesure où elle permet à chacune et à chacun de développer son esprit critique. C'est la grande utilité du service public que d'apporter ces instruments de la critique à tout le monde. Il n'est pas suffisamment dit que ces actions, loin d'être rébarbatives, suscitent l'adhésion franche du public. Sans être injuste, j'aimerais citer l'exemple de France Culture, dont les audiences ont fortement augmenté grâce à une politique de contenus exigeante. Parmi ces productions, il faut citer le développement exceptionnel de la diffusion des contenus sur internet. Je crois que ces succès ne sont pas assez connus ni assez mis en valeur. Il serait souhaitable que tous ces contenus soient valorisés sur un portail dédié et plus facilement accessible. Je pense notamment à tous ces- balados, -téléchargés à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires qui mériteraient d'être mieux diffusés par le biais d'applications plus adaptées et plus accessibles. Le service public de l'audiovisuel a besoin d'un plan d'investissement massif pour adapter toutes ces pratiques à l'internet. La

interrogerai ensuite sur votre vision du rayonnement de notre audiovisuel extérieur. Force est de reconnaître que, en à peine treize ans d'existence, France 24 a su faire entendre une voix originale aux côtés de concurrents aussi importants que CNN, BBC World News ou Al Jazeera. Cette voix porte les valeurs de la France et décrypte le monde à travers elles. Pour porter cette ambition, France 24 mérite mieux. Elle aurait d'ailleurs pu être le socle de lancement de la chaîne d'information française qui a eu le mérite de rassembler France Télévisions et Radio France.

car l'audiovisuel extérieur est un relais capital du rayonnement international de la France. Il a vocation à porter une vision française de l'actualité sur la scène internationale et à promouvoir la francophonie, sujet qui nous tient à coeur, vous le savez. Pour accompagner cette mission

de 2,5 %, soit la plus forte hausse de toutes les entreprises de l'audiovisuel public pour 2018. J'ai ainsi entendu poursuivre l'effort important de soutien à l'audiovisuel extérieur engagé par l'État depuis cinq ans. Entre 2013 et 2017, sa dotation a en effet

L'audiovisuel public extérieur doit aussi bénéficier de coopérations accrues avec l'ensemble des sociétés audiovisuelles. Il existe ainsi des coopérations entre Arte et France 24 sur l'offre hispanophone. D'autres partenariats sont en cours et s'établissent au fur au fur et à mesure des comités stratégiques. J'ai lancé un chantier de réflexion dans ce cadre-là.

Les réformettes, c'est fini pour le service public. Il faut cette fois-ci avoir une grande ambition. Il faut permettre d'opérer des synergies. » Cette phrase ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été prononcée non par vous, madame la ministre, mais par Hervé Bourges, alors président d'Antenne 2 et de FR3, en 1991. Elle témoigne, s'il en était besoin, que la réforme de l'audiovisuel public est un chantier aussi ancien que périlleux. Cette réforme revêt cependant un caractère d'urgence alors que la révolution numérique bouleverse les usages et les rapports aux contenus audiovisuels de bon nombre de nos concitoyens.

financement de l'audiovisuel public, procédure de nomination de ses dirigeants et, surtout, réorganisation fonctionnelle et refonte de l'offre de programmes. Ma question porte spécifiquement sur le chantier de l'amélioration de l'offre de proximité et concerne plutôt les réseaux France Bleu et France 3, lesquels ont déjà connu une réorganisation afin de leur permettre de s'adapter au nouveau cadre institutionnel des grandes régions. Une communication de proximité est souhaitable, et souhaitée, par les élus et les téléspectateurs, pour permettre à chacun de s'approprier le nouveau périmètre régional, mais aussi pour conserver et renforcer la notion d'identité locale. Il est question de rapprochement- immobilier, mais pas seulement -et de programmes en commun, notamment lors de la tranche matinale. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, les arbitrages qui ont été faits sur les préconisations qui vous ont été adressées et sur le calendrier des prochaines échéances ? Plus largement, pouvez-vous nous éclairer sur votre vision, votre cap, s'agissant d'un renforcement de l'audiovisuel public de proximité et de qualité,

Vous le savez, l'offre de proximité remplit des missions essentielles pour la cohésion sociale au plus près des territoires, la mise en valeur des événements culturels régionaux et la démocratie locale.

typiquement le genre d'offre qui n'est pas fournie par les chaînes privées ou par les GAFAN. C'est la spécificité du service public, qui doit jouer pleinement son rôle.

Chez France Bleu, on trouve des gens d'une grande agilité, qui ont envie de travailler et d'être complémentaires. Des coopérations peuvent se mettre en place, comme cela s'est passé à l'échelon national avec France Info.

Gallet, premier PDG à avoir été révoqué pendant son mandat. Cette décision prendra effet le 1 mars prochain. Le rapport des sénateurs Gattolin et Leleux de 2015 explicite les problèmes soulevés par la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le CSA. pour l'élection présidentielle, le président Macron a repris ses conclusions et a affirmé vouloir en finir avec ce mode de désignation. Or l'idée de changer rapidement la règle par le vote d'une petite » loi a été abandonnée. C'est donc bien le CSA qui nommera le successeur de M. Gallet, au terme d'un processus de candidature, d'auditions et de vote s'étalant sur deux mois et demi environ.

Mme la ministre.

Dans l'attente de la nomination d'un nouveau président, c'est le doyen des administrateurs, M. Jean-Luc Vergne, qui assure la transition. Ce qui est important, c'est que Radio France continue. Les équipes sont au travail.

Le mode de financement actuel de l'audiovisuel n'est plus adapté, nous le savons. La publicité, en particulier, ne fait plus recette à la télévision. La bascule des budgets publicitaires entre la télévision et internet a eu lieu plus tôt que prévu. Initialement attendue pour 2018, elle s'est en fait

Doit-il y avoir de la publicité sur les chaînes du service public ? Progressivement, nous sommes allés vers sa suppression. Depuis 2009, il n'y a plus de publicité après vingt heures sur les chaînes de France Télévisions. Le Sénat, vous le savez, a été en pointe pour étendre cette suppression. C'est en effet une proposition de loi sénatoriale qui a supprimé la publicité dans les programmes pour la jeunesse de la télévision publique. Pourtant, le débat est loin d'être tranché. Certains plaident pour le retour de la publicité le soir sur France Télévisions. À l'inverse, des dirigeants de chaînes privées réclament la suppression totale de la publicité sur le service public. Madame la ministre, quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet ? Quel est le bilan de la suppression partielle de la publicité sur France Télévisions ? Le retour de la publicité heures est-il envisageable ? Au contraire, va-t-on vers une suppression complète de la publicité sur France Télévisions ?

En 2017, France Médias Monde a confirmé ses bons résultats d'audience, notamment en Afrique francophone où France 24 est la première chaîne d'information internationale et RFI, de très loin, la première radio internationale. Le lancement de France 24 en espagnol en septembre 2017 montre également l'expansion de ce média à l'international. Ces beaux succès sont dus au formidable travail et à l'engagement des équipes dirigées par Marie-Christine Saragosse. Si des synergies sont indispensables, comme l'a montré récemment le lancement de la nouvelle chaîne publique France Info TV, France Médias Monde et TV5 Monde, médias francophones, possèdent, par leur histoire et leur financement, une identité propre. À l'heure où le Président de la République a fait de la francophonie une priorité, nous devons montrer notre attachement à l'audiovisuel extérieur, qui est l'une de ses plus belles vitrines. Madame la ministre, la présidence commune aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde envisagée par le Gouvernement ne risque-t-elle pas de constituer un frein au développement de l'audiovisuel extérieur, dont les missions très spécifiques peuvent difficilement être assujetties aux problématiques de l'audiovisuel national

pauvre de la politique audiovisuelle française. Il ne représente en effet que 7 % de son budget. Or l'audiovisuel extérieur, incarné par France Médias Monde, est un levier

en tête, font des médias un majeur pour étendre leur influence, la France ne peut pas se permettre d'affaiblir son audiovisuel extérieur. Le Président de la République souhaite procéder à une réforme afin de rapprocher les sociétés de l'audiovisuel public, d'en mutualiser la gouvernance et d'en améliorer l'efficacité. Le

cette façon d'envisager la gouvernance ne remet absolument pas en cause l'importance et les spécificités qu'il s'agit d'attacher à chaque secteur de l'audiovisuel public, tout particulièrement celui

en particulier celui de France 3 et de France Bleu. Cette coopération renforcée s'accompagnerait d'une fermeture des bureaux régionaux de France 2 et d'un recentrage de l'offre régionale de France 3. Or l'information de proximité est bien le coeur de mission de de France 3. À la fin de 2017, les antennes locales de France 3 se sont émues de l'annonce de l'arrêt de leur diffusion à compter du 1 janvier 2018. La direction régionale de France 3 Bretagne avait alors souligné que la réflexion en cours avait pour objectif de maintenir la production des contenus au niveau local par des journalistes sur le terrain, dont la liberté de ton est spécifique à France 3, et de les diffuser sur internet ainsi que sur les antennes régionales, pour atteindre un public plus large. Cette évolution devrait permettre de rendre plus visible le travail des journalistes locaux, en variant les supports de diffusion. Une telle décision va dans le sens du rapport rendu en 2014 par la mission menée par Anne Brucy, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. La mission y mettait en évidence l'atout que constitue la télévision régionale et locale et soulignait déjà la nécessité d'en adapter la diffusion aux nouvelles technologies. Mais, de ce rapport, En Bretagne, France 3 coopère déjà avec le réseau France Bleu pour couvrir des événements sportifs et culturels importants. Il s'agit cependant non pas d'une expérimentation à proprement parler, mais d'une collaboration Madame la ministre, vous affichez à la fois une ambition pour un service public de qualité et un attachement à une offre d'information de proximité dans les territoires. Dès lors, en quoi consistera exactement le rapprochement entre ces deux réseaux, et quel en sera l'impact ?

depuis plusieurs mois, notamment depuis le vote du budget pour 2018, l'avenir de l'audiovisuel public fait l'objet de toutes les attentions et de moult commentaires, y compris au plus haut niveau de l'État. Il faut dire que cette question est loin d'être neutre tant les enjeux sont importants et les conséquences bien réelles. C'est pourquoi je me réjouis que nous puissions aborder ce sujet ce soir au sein de notre Haute Assemblée, car, effectivement, le mode de gouvernance et les outils de l'audiovisuel français ne paraissent plus adaptés à la réalité. Tout d'abord, parlons de son financement. Avec une redevance fixée à 138 euros par an, la France se situe dans la fourchette basse par rapport à nos voisins puisque, en Grande-Bretagne, elle s'élève à 202 euros, en Allemagne, à 216 euros, et en Suisse, à 316 euros. Nos amis helvètes vont d'ailleurs se prononcer le 4 mars prochain lors d'une votation sur le bien-fondé de ladite taxe qui finance des chaînes publiques. Ces chaînes linéaires ne sont pas regardées par tous les Suisses, puisque nombre d'entre eux, notamment les plus jeunes, sont abonnés à des chaînes privées. C'est bien là l'enjeu. Car ce qui pouvait apparaître comme une forme de solidarité territoriale voilà encore quelques années, avec l'objectif d'implanter France 3 dans les régions, n'est plus le reflet de la réalité d'aujourd'hui. D'ailleurs, cette représentation territoriale a-t-elle été seulement effective ? Dans les territoires ruraux, peu peuplés, nous ne pouvons pas dire que nous ayons bénéficié un jour d'un service audiovisuel public qualitatif, représentatif de notre spécificité. Par exemple, mon département, celui des Hautes-Alpes, n'a jamais été couvert par le réseau France Bleu. Actuellement se pose en effet la double question de la répartition financière et de l'absence de péréquation au bénéfice des départements peu peuplés, ainsi que de la qualité et du pluralisme des programmes indépendamment des critères de rentabilité. C'est pourquoi, madame la ministre, dans le cadre de la réforme qui pourrait intervenir, je vous demande de préciser les mesures envisagées pour corriger la fracture territoriale dans l'audiovisuel public. La parole est à Mme la ministre.

Afin de garantir un aménagement harmonieux du territoire lors du passage à la télévision numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est assuré que la couverture numérique de chaque département serait égale ou supérieure à la couverture analogique. Pour les téléspectateurs situés en zone blanche de la TNT, que vous évoquez, la loi a prévu un accès à l'ensemble des chaînes par satellite sans abonnement. Ce dispositif complémentaire garantit à l'ensemble des foyers un accès gratuit aux 27 chaînes de la TNT, la plupart en haute définition.

objectifs : la reconquête des jeunes, la gouvernance, la mutation numérique, le renforcement de la culture. Si nous pouvons partager ces ambitions, je regrette à titre personnel, au moment où nos athlètes font briller les couleurs de la France en Corée du Sud, que la diffusion des compétitions sportives ne

et, surtout, sur les moyens qui y seront dédiés dans la perspective de l'accueil des grandes compétitions internationales, notamment des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Aujourd'hui, les tractations sur l'acquisition des droits audiovisuels des Jeux de 2024 sont en cours. Plus que jamais, c'est un défi pour la France, pour France Télévisions, alors que Discovery France a annoncé que ces droits seraient au moins aussi chers que pour un Mondial de football. La diffusion des Jeux, des compétitions sportives en général, permet de véhiculer des messages de santé publique.

Le CSA, dans une note publiée la semaine dernière, considère qu'une amélioration est à envisager pour retransmettre encore plus d'épreuves en 2024 sur France Télévisions. Dans le cadre de la rénovation de l'audiovisuel public, madame la ministre, le Gouvernement est-il prêt à à soutenir pleinement, et donc financièrement, France Télévisions et sa politique en faveur du sport, afin de permettre une très large diffusion de l'ensemble des épreuves et des disciplines des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ? Plus largement, quelle place aura le sport dans ce renouveau de l'audiovisuel public ?

est un événement national extrêmement fédérateur, que tous les Français doivent pouvoir vivre et partager. Je souhaite donc effectivement une large ouverture des jeux Olympiques de Paris sur les chaînes gratuites. C'est d'ailleurs pour cette raison que la compétition est un événement d'importance majeure au regard de la réglementation française. Ce sujet est bien connu de votre collègue David Assouline, qui a rendu un rapport à ce sujet. Les JO sont une compétition la présence de tout ou partie des épreuves sportives sur les antennes du service public est donc légitimement attendue. Pour autant, au regard du contexte économique de l'audiovisuel public, nous devons veiller à ce que l'acquisition de ces droits de diffusion ne soit pas réalisée à n'importe quel prix. Des discussions sont